avons terminé avec le débat sur le thème « La caducité du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne rendra-t-elle une autonomie budgétaire aux États membres ? » Mes chers collègues,

La réforme de la zone euro est à nouveau à l'ordre du jour. Parmi les pistes envisagées, l'évolution des règles budgétaires devrait figurer en tête de liste. Celles-ci ont en effet engendré une austérité budgétaire excessive pendant la crise, aggravant et prolongeant ses conséquences économiques, sociales et politiques Ces règles souffrent en outre de graves problèmes de mesure : elles sont basées sur un concept légitime, le solde public structurel, mais celui-ci n'est pas observable et fait l'objet d'importantes erreurs d'estimation Ces quelques lignes, mes chers collègues, n'émanent pas d'une analyse du parti communiste. Non, cette prise de position est celle du Conseil d'analyse économique ! Elle nous appelle clairement, plus de vingt-cinq années après le traité de Maastricht, plus de dix ans après l'explosion de la profonde crise du capitalisme en 2007, à remettre en cause l'inefficacité et l'injustice de l'encadrement des politiques budgétaires nationales.

Cet événement essentiel est pourtant étonnamment passé sous silence par notre gouvernement, alors même que nous sommes en pleines élections européennes et que l'injustice fiscale et les conséquences de l'austérité sont largement mises en cause dans notre pays. Dans tout l'arsenal « austéritaire » mis en place par les gouvernements à l'échelle européenne, le TSCG, signé en 2012, tient une place particulière. Résultat de la collaboration entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, il fut au coeur de la campagne présidentielle de 2012 et, malgré les promesses de renégociation faites par François Hollande devant les Français, il fut signé sans qu'une ligne Nous avions dénoncé ce déni de démocratie, ainsi que les dangers de ce corset budgétaire, et démontré à l'époque au Parlement européen les problèmes de légalité posés par ce traité. En effet, le TSCG poussait comme jamais à l'encadrement et au contrôle constitutionnel ou quasi constitutionnel de l'action publique et budgétaire des gouvernements nationaux. En cela, il s'oppose frontalement à la tradition républicaine d'une souveraineté parlementaire sur les dépenses de la Nation. Des mécanismes de contrainte de la dépense publique avaient déjà été imposés avec les règlements et. Mais le TSCG porte, lui, une atteinte inédite à la souveraineté, au travers de trois éléments centraux son article 3 introduit la règle d'or, au travers du respect d'un déficit structurel de l'État membre ne dépassant pas l'objectif à moyen terme qui lui est propre, dans la limite de 0,5 % du PIB deuxièmement, la soumission à des recommandations du Conseil européen et, au titre de l'article 7 du TSCG, l'établissement d'une majorité qualifiée inversée au Conseil pour échapper à ces recommandations la soumission du contrôle de ces recommandations dans les budgets nationaux à la Commission européenne. Aujourd'hui, les conséquences de ces politiques d'austérité sont connues ; elles sont dramatiques. Elles ont signé l'abandon de toute ambition de politique publique en Europe, pourtant si nécessaire à la réduction des inégalités, comme à la conduite de long terme des indispensables transitions industrielles et écologiques.

La bête noire de nationalismes xénophobes resurgit dans toute l'Europe, et l'abstention s'annonce comme la grande gagnante des élections européennes à venir. Dans l'Europe des années 1930, le philosophe Edmond Husserl le disait déjà Le plus grand danger pour l'Europe est la lassitude. » En 2019, il s'agit de la lassitude face aux mécanismes d'austérité, mais aussi face à un avenir sans cesse plus obstrué. Nous ne nous résignons pas à cette dangereuse lassitude. Nous proposons donc de nous saisir d'une situation exceptionnelle dans l'édifice juridique européen : la caducité avérée du TSCG. La vérité doit être dite aux Français : depuis décembre 2018, soit moins de six mois, la France et les autres États européens ne sont plus liés par les dispositions du TSCG. La règle d'or, le mécanisme de majorité inversée et la soumission des budgets à la Commission ne sauraient plus constituer des obligations juridiques s'imposant aux États membres de la zone euro. Je veux prouver ce que nous affirmons, car nous savons que les dogmatiques de l'austérité vont s'accrocher à ces politiques pourtant partout rejetées en Europe. Tout d'abord, le TSCG n'est pas un traité de droit européen et ne l'a jamais été. À l'image du mécanisme européen de stabilité, il constitue un outil de droit international, soumis, par conséquent, aux règles coutumières de ce dernier. Si le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est, au titre au titre de son article 356, conclu pour une durée illimitée, tel n'est pas le cas du TSCG, traité « temporaire » dont le caractère transitoire découle de son article 16, qui fixe un délai de cinq ans maximum pour sa transposition en droit européen. Or ce délai est épuisé, et il n'y a pas eu de transposition. Dans la proposition de directive soumise en décembre 2018 par la Commission, le caractère transitoire est rappelé avec clarté : « Les parties contractantes ont exprimé leur volonté d'utiliser cet instrument intergouvernemental comme dispositif temporaire. Cette volonté est reflétée à l'article 16 du TSCG, qui prévoit que, « dans un délai de cinq ans maximum à compter de la date d'entrée en vigueur dudit traité, les mesures nécessaires sont prises afin d'intégrer le contenu du traité dans le cadre juridique de l'Union européenne. » Ce caractère transitoire a aussi été remarqué par le Conseil constitutionnel français. Dans le propre commentaire de leur décision 2012-653 DC relative au TSCG, les Sages déclaraient ainsi clairement : « Ce traité a une vocation transitoire. Or, si en vertu de l'article 55 de notre Constitution, les engagements internationaux ratifiés et approuvés sont applicables et supérieurs aux lois, la jurisprudence a, à de nombreuses reprises, souligné qu'une telle situation ne trouvait à s'appliquer que dans la mesure où ces engagements étaient régulièrement ratifiés et toujours en vigueur. La situation de caducité du TSCG est donc clairement établie. Au terme des cinq ans, la commission des affaires économiques du Parlement européen s'est opposée à la proposition de directive de la Commission européenne transposant le TSCG en droit européen ; il s'agit clairement, dans la procédure législative européenne, d'un refus, qui, normalement, doit mettre un terme au projet de la Commission. Du point de vue du droit international, la situation est claire : dans le cas de traités conclus pour une durée déterminée, ceux-ci cessent d'être applicables dès qu'ils sont arrivés à expiration, sans qu'une dénonciation soit nécessaire. J'entends l'autre objection que vous pourriez nous opposer : une loi organique ayant été votée en France, le droit interne suffirait donc à soumettre les budgets nationaux à la règle d'or. C'est oublier deux choses essentielles. part, l'enjeu de la caducité du TSCG dépasse les seules frontières nationales et engage l'ensemble de l'Europe. D'autre part, la transposition du TSCG en France ne s'est pas faite- c'est le moins que l'on puisse dire -sans réticence des parlementaires ou des juges nationaux. Il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle, et le déficit structurel de 0,5 % du PIB n'a pas été inscrit,, dans la loi organique. Dans ce cadre, aucune disposition constitutionnelle ne saurait plus nous obliger à respecter un objectif de moyen terme de 0,5 % de déficit structurel. Une telle position est, par ailleurs, en cohérence avec l'avis formulé par le Conseil d'État relatif à la loi de programmation 2009-2011. Mes chers collègues, avec la caducité du TSCG en Europe, c'est l'un des mécanismes structurants de la conception de l'encadrement des politiques publiques qui est mis en cause. En France, c'est la conception qui préside aux lois de finances pluriannuelles qui est contestée. Alors que nos citoyens, nos travailleurs, nos PME, nos agriculteurs, nos artisans, nos services publics sont étranglés par les politiques d'austérité, nous devons saisir cette occasion historique. La France doit prendre la tête du combat pour libérer l'Europe des mécanismes de contrainte, qui ont étouffé l'activité économique, enrichi les actionnaires et appauvri les peuples et les nations. L'Europe fait face à des défis cruciaux, industriels, économiques, informationnels. Ces derniers ne pourront être atteints sans l'engagement de la puissance publique, sans de réels mécanismes de coopération budgétaire en Europe. J'ai rappelé ici il y a quelques jours, en présence du ministre Bruno Le Maire, nos propositions pour la création d'un fonds de développement des services publics et pour la refondation des missions de la Banque centrale européenne au service d'un nouveau développement social, industriel et écologique. Le vide juridique laissé par la caducité du TSCG doit nous libérer des multiples instruments de contrainte budgétaire qui ont violé les souverainetés nationales en Europe. D'autres traités de droit international peuvent être négociés pour, enfin, mettre sur rail une nouvelle union des peuples et des nations libres, souverains et associés. Mes chers collègues, déjà en son temps Voltaire s'interrogeait : « La vieille Europe, elle ne revivra jamais ; la jeune Europe offre-t-elle plus de chances ? À l'approche de ces élections européennes, qui se révèlent cruciales pour l'avenir de notre continent, donnons enfin une réponse qui soit à la hauteur des enjeux que nous affrontons dans notre époque. La

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, notre groupe a souhaité porter à l'ordre du jour de notre assemblée la question de la caducité du TSCG. Notre collègue Pierre Laurent vient de démontrer avec force arguments combien la France ne devait plus être liée par les dispositions contenues dans ce traité. Dans le prolongement de cette première intervention, je voudrais souligner la nécessité pour la France et pour l'Europe de rompre, de manière durable, avec la logique même portée par le TSCG et les autres règles d'encadrement budgétaire européen. Caduc juridiquement, ce traité, ainsi que l'ensemble des règles européennes contraignantes des politiques budgétaires, est également dépassé économiquement, socialement et politiquement. Ils ont fait la preuve de leur inefficacité ainsi que de leur injustice. Économiquement, tout d'abord, les prémisses théoriques des instruments actuels du contrôle budgétaire postulent l'inefficacité de la dépense publique et conduisent, en définitive, à faire primer la libre action des acteurs privés sur les marchés. De plus, le Conseil d'analyse économique, que Pierre Laurent a cité, critiquait dans une note de septembre 2018 la mesure du solde structurel qui, pourtant, sert de base au fonctionnement du TSCG et des autres mécanismes de contrôle budgétaire.

L'Europe en paye aujourd'hui les conséquences. C'est particulièrement vrai dans les industries et les secteurs de pointe, où la production européenne est en grand recul. À titre d'exemple, la part de l'industrie dans le PIB européen est passée au-dessous des 20 %, quand elle dépasse en Chine les 40 %. Pis encore, les règles européennes d'encadrement des finances publiques sont aujourd'hui contraires aux maigres volontés d'investissement des gouvernements européens, à l'image du plan que le ministre allemand Peter Altmaier a présenté la semaine passée. Ces règles étaient un handicap ; elles se transforment aujourd'hui en obstacle. Même les dirigeants allemands de la CDU-CSU commencent à en prendre conscience. Ces règles étaient restrictives, elles sont aujourd'hui dépassées dans la compétition mondiale. Elles empêchent, dans les faits, de mener des stratégies ambitieuses pour nos entreprises, les PME, nos artisans et, surtout, nos territoires. L'insistance des règles européennes à faire respecter une trajectoire de solde structurel vers 0,5 % est également dépassée socialement. Le TSCG, les dispositions du traité de Lisbonne, les et empêchent les États membres de mener des politiques de cohésion sociale adaptées aux besoins des populations. Réduire, arbitrairement, les moyens de l'action publique dans des temps de crise conduit 87 millions d'Européens à survivre sous le seuil de pauvreté. Surtout, ces politiques font porter sur les épaules des plus fragiles le fardeau de l'économie financiarisée et de ses crises à répétition. L'inclusion dans les règles du TSCG et les autres mécanismes européens de toutes les dépenses des administrations publiques, sociales, militaires, économiques, sans aucune pondération particulière, est également injuste socialement. Elle empêche toute protection privilégiée des dépenses sociales, alors même que celles-ci sont, dans les temps de crise, indispensables pour maintenir la cohésion de nos sociétés. Politiquement, enfin, les règles actuelles contraignent la souveraineté des parlements européens. Elles participent directement à la mise à distance des peuples de la construction européenne. Elles contribuent aussi directement à la montée des forces nationalistes, qui, de l'Espagne à la Hongrie, de l'Estonie à l'Italie, favorise les courants les plus réactionnaires. Il est l'heure de proposer, à l'occasion des prochaines élections européennes, un nouvel horizon pour nos finances publiques, en France et en Europe. En France, libérés de l'objectif de solde structurel à l'horizon de 2022, nous pourrions désormais planifier un autre chemin de développement, protecteur des plus fragiles et redonnant de l'air à nos entreprises. Notre vision des finances publiques s'articule autour de deux piliers : la justice sociale et territoriale, d'une part ; l'efficacité économique, d'autre part. La justice sociale et territoriale, tout d'abord. Plus que la contrainte et la négation de la libre administration des collectivités territoriales, nous pouvons en finir avec la contractualisation qui a été pensée et appliquée dans l'objectif du respect du solde structurel. Les dépenses de cohésion sociale, le soutien aux administrations de sécurité sociale devraient être considérés comme prioritaires, et, à l'inverse, il faut en finir avec l'impulsion donnée aux dépenses militaires. Mes chers collègues, une gestion socialement juste est une affaire de choix avant tout. Entre la dépense militaire et la dépense hospitalière, nous assumons pleinement les nôtres. La justice doit également primer dans les recettes de l'État. À ce titre, nous voulons, une fois encore, réitérer nos positions de principe, qui sont très largement partagées dans la population. Ainsi, nous voulons le rétablissement de l'impôt et de l'imposition progressive sur le capital, de même qu'une refonte des tranches de l'impôt, pour atteindre, à terme, quatorze tranches d'impôt sur le revenu. Nous voulons, ensuite, favoriser l'efficacité économique. Là encore, la logique du TSCG et la volonté purement comptable de tenir l'objectif de moyen terme ont été largement négatives pour notre économie. Nous souhaitons une refonte du soutien public à nos entreprises, une pérennisation de nos fleurons industriels, un fonds d'investissement social et écologique pleinement actif. Enfin, mes chers collègues, c'est l'Europe qui doit prendre un tout autre chemin. La contrainte budgétaire anachronique pèse fortement sur l'avenir de notre continent. Libérée de la logique du TSCG, l'Europe doit pouvoir se ressaisir, adopter une politique réaliste dans son soutien à l'activité, faire primer les logiques productives et sociales plutôt que le libre-échange généralisé. La parole Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il n'est pas possible d'avoir durablement une monnaie commune sans une politique budgétaire et monétaire commune ou, au moins, convergente. Et dans un espace de libre circulation, la convergence budgétaire ne peut se faire sans convergence fiscale. Les créateurs de l'euro, je le pense, n'ignoraient pas cette évidence,

tenu. En 1997, le pacte de stabilité et de croissance a mis en place une sorte de pilotage automatique des politiques budgétaires des pays qui allaient faire partie de la zone euro. En 2008, la crise a mis en danger l'ensemble de l'édifice, et il a fallu revoir les choses dans l'urgence, tant s'agissant de la convergence budgétaire qu'en termes monétaires. Le premier pas, douloureux,

De fait, la politique de concurrence européenne est aussi devenue caduque parce que le marché européen n'a pas été suffisamment soutenu. La réduction du périmètre de l'action publique dans les différents pays européens,

il n'était donc pas du tout raisonnable, comme le proposait le parti populaire européen, d'inscrire les dispositifs du TSCG dans les traités de l'Union européenne.

une réponse adéquate pour une politique budgétaire plus intégrée entre les pays de la zone euro. Le pacte de stabilité lui-même doit être revu.

Enfin, c'est bien parce que nous voulons que l'Europe soit un modèle pour l'avenir, en particulier pour la transition énergétique, qu'il est absolument indispensable de renforcer les capacités d'endettement de la puissance publique.

Ce manque d'investissements en Europe est particulièrement dramatique au regard de ce qui se passe dans d'autres pays- je reviens de Chine. Ne nous trompons pas sur Donald Trump, qui, dans son pays, augmente de manière importante

de démocratisation de l'Europe permettrait de les remettre au coeur des décisions européennes et des choix économiques et sociaux qui doivent être faits. Il ne faut pas attendre la prochaine crise pour agir,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce débat, organisé sur l'initiative de nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, mériterait sans doute plus qu'une heure, compte tenu de tout ce qui a déjà été écrit ou dit sur les critères européens et des discussions qu'ils continuent de susciter. ne se limitent d'ailleurs pas au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de 2012, qui n'est que le dernier étage d'un ensemble de règles instaurées avec les traités de Maastricht en 1992, puis d'Amsterdam en 1997, à l'origine du pacte de stabilité et de croissance.

règle a ensuite été reprise lors des négociations du traité de Maastricht et de l'instauration de l'Union économique et monétaire. Il faut donc inverser la vision commune de cette règle des 3 % : ce n'est pas l'Europe qui aurait imposé une règle budgétaire arbitraire aux États membres celle-ci a été introduite dans les traités sur l'initiative de la France, avec l'accord de l'Allemagne, qui souhaitait garantir une certaine discipline budgétaire au sein de l'Union. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne, adopté en 2012-2013 dans les conditions que l'on sait, n'a fait que renforcer ou affiner ces règles, en introduisant la notion de solde structurel et l'objectif de moyen terme, que nous avons adopté en loi de programmation, en fixant un objectif de réduction de la dette d'un vingtième par an- le « pacte budgétaire » -et en renforçant la coordination des politiques économiques et la gouvernance de la zone euro. Aujourd'hui, force est de constater que, depuis l'origine, aussi bien le pacte de stabilité et de croissance que le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance ont été relativement peu respectés par les États membres, en particulier par la France, qui, hélas, ne figure pas parmi les bons élèves. En effet, notre pays présente encore un déficit structurel supérieur à 0,5 point de PIB, même s'il existe des débats d'experts sur la délimitation exacte de ce qui relève respectivement du conjoncturel et du structurel, voire de l'exceptionnel. Ainsi, sur 2019,

à l'année budgétaire. La crise financière de 2008 et la crise des dettes publiques ont porté le coup le plus sévère aux règles du pacte de stabilité. De nombreux États qui avaient redressé la barre ont dû recourir à des déficits très supérieurs à 3 %. Cela a entraîné une hausse spectaculaire de l'endettement public : alors que la France était en 2008 tout juste dans la limite des 60 % d'endettement, elle approche désormais des 100 %, avec toutefois une stabilisation depuis 2017. La situation des déficits s'est améliorée. En 2018, seule l'Espagne affichait un déficit encore supérieur à 3 %, et quatorze pays, dont la Grèce, présentaient un budget en équilibre ou en excédent. Depuis 2017, la France a un déficit inférieur à 3 % du PIB et elle est enfin sortie de la procédure de déficit excessif. En revanche, le niveau d'endettement reste élevé : la moitié des États membres présentent une dette publique supérieure à 60 %, et cinq pays ont une dette supérieure à 100 % du PIB. La dette moyenne dans la zone euro était de 86 % en 2018. Nombreux sont ceux qui, depuis l'origine ou plus récemment, remettent en question les critères de convergence européens. De fait, au niveau de l'Union, la France, qui porte depuis longtemps le projet d'une Union économique et politique plus étroite, avec une véritable gouvernance de la zone euro et un budget commun, doit composer avec les réticences de l'Allemagne et d'autres États, qui craignent de devoir payer pour la mauvaise gestion réelle ou supposée de leurs voisins. Alors que le fédéralisme est aujourd'hui très poussé en matière monétaire, et qu'il s'est renforcé dans le domaine bancaire, la politique budgétaire reste le parent pauvre ce qui laisse le système européen incomplet et déséquilibré. Dans ce contexte, qu'apporterait réellement une sortie des traités ? La situation outre-Manche est éclairante à cet égard. Au-delà des négociations difficiles sur le Brexit, le Royaume-Uni offre l'exemple d'un État membre qui n'a pas signé le Pacte budgétaire

dû mettre en place leurs propres règles contraignantes, afin de maîtriser leurs finances publiques. Depuis de nombreuses années maintenant, ils pratiquent une austérité budgétaire qui n'aurait probablement pas de quoi enchanter nos collègues. Brexit ou pas à la fin de l'année, il n'est pas sûr qu'ils y mettent un terme dans un avenir proche. Cet exemple semble donc indiquer qu'une sortie pure et simple des traités ne ferait pas disparaître certaines contraintes qui s'exercent sur nos finances. Enfin, il faut rappeler le contexte de l'adoption du Pacte budgétaire. C'était alors la condition qu'avaient posée l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres pays pour poursuivre l'aide aux pays en difficulté financière, en particulier la Grèce. La volonté d'apporter une réponse aux causes structurelles des déficits n'est pas critiquable en soi, me semble-t-il. En revanche, la question de la convergence continue de se poser. L'absence de politique budgétaire proprement européenne reste un frein à une véritable coordination et à une politique plus tournée vers l'investissement, la croissance, l'emploi et la transition énergétique, ce à quoi devait répondre le Pacte pour la croissance de 2012. C'est le sens de la proposition réitérée par le Président de la République à nos partenaires européens. Le rôle des parlements nationaux, tel qu'il est défini aux articles 3 et 13 du traité, mériterait également davantage d'attention. Ces quelques remarques montrent la complexité du sujet. Il est improbable qu'une sortie sèche des traités fasse disparaître les contraintes qui pèsent sur la politique budgétaire des États membres. En revanche, la zone euro doit mettre beaucoup plus l'accent sur l'investissement, l'emploi et la coordination budgétaire et fiscale. conclure, si cette règle des 3 % qui nous est imposée par l'Europe - il est facile de renvoyer l'impopularité de telles contraintes sur d'autres d'autres ! -n'existait pas, nous devrions nous l'imposer à nous-mêmes. L'objectif est non pas de se limiter à la règle des 3 %, mais d'avoir un budget en équilibre et même, si possible, excédentaire, afin d'amorcer la réduction de l'endettement public. Notre surendettement nous prive aujourd'hui de toute marge de manoeuvre. Il affaiblit politiquement notre pays, en nous privant des moyens financiers qu'il serait souhaitable de mobiliser pour la modernisation de nos infrastructures routières, ferroviaires, fluviales ou hospitalières, pour la transition énergétique ou encore pour l'aide au développement en faveur, par exemple, des pays africains. Il faut conclure, mon cher collègue. L'absence de contraintes budgétaires est synonyme non pas d'autonomie budgétaire, mais plutôt d'impuissance politique.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, alors que nous célébrons aujourd'hui la journée de l'Europe, je remercie nos collègues du groupe CRCE d'avoir fait inscrire ce grand et beau projet qu'est le projet européen à l'ordre du jour de notre assemblée. Cependant, quel paradoxe de polariser le débat sur la gouvernance de la zone euro

Cette critique, mes chers collègues, vous ne pouvez pas nous empêcher de penser qu'elle est motivée autant par une forme de nostalgie que par une volonté de justice sociale ou territoriale. Quel dommage que votre vision de l'Union européenne soit ainsi centrée sur les contraintes, les seules contraintes qu'elle imposerait aux États ! Mettons tout d'abord les choses au clair : malgré ce que l'on peut lire dans une certaine presse, le traité de stabilité dont il est question aujourd'hui n'est pas caduc. Si, il l'est ! Le retard pris, il est vrai, par rapport aux dispositions de son article 16, ne saurait en entraîner la caducité. Toujours en vigueur, il mérite tout notre sérieux. Le contenu et la philosophie de ce traité placent de fait la discipline budgétaire en son coeur. Cependant, et de manière cohérente avec l'esprit des règles européennes, elle s'accompagne de deux autres piliers tout aussi importants : la coordination des politiques économiques des États membres et la gouvernance de la zone euro. Ces trois composantes ne sauraient aller l'une sans les autres, au risque de déséquilibrer l'approche même de l'Union européenne sur ce sujet. Les dispositions relatives à la discipline budgétaire énoncent en effet des règles complémentaires à celles du pacte de stabilité et de croissance pour les pays de la zone euro. Je n'entrerai pas ici dans le détail des mesures techniques, ce qui a déjà été fait, mais je ne puis qu'insister sur le fait que de telles dispositions sont aujourd'hui encore nécessaires au bon fonctionnement de l'espace économique commun et intégré qu'est l'Union européenne. L'établissement, pour chaque pays, d'un objectif de réduction de sa dette devient alors un gage de pérennité pour l'ensemble du système, la crise grecque ayant démontré le danger que peut représenter le risque de défaut d'un seul État. Par ailleurs, notons que le traité introduit une évolution intéressante avec le choix d'évaluer le déficit structurel des États membres. Cela permet de mieux prendre en compte l'impact d'une crise économique que l'étude du seul déficit public tant décrié. Le traité organise par ailleurs une coordination accrue des politiques économiques des États membres. Si cette approche était essentielle au moment de la signature du texte en 2012, elle ne l'est pas moins en 2019, pour les pays membres de la zone euro comme pour l'ensemble de l'Union. En effet, le traité engage notamment les États membres à débattre préalablement de leurs mesures économiques domestiques et à les coordonner au maximum. Cela peut paraître évident, mais il est toujours bon de rappeler que l'Union européenne ne pourra faire face aux grands blocs économiques que sont les États-Unis et la Chine qu'en abordant les grands enjeux du moment d'une seule voix. La coordination est, à cet égard, plus que jamais nécessaire. Enfin, la gouvernance de la zone euro s'est trouvée renforcée par ce traité grâce à l'institution des sommets de la zone euro, ainsi que par une association plus étroite des parlements nationaux au débat économique européen. Les marges de progrès existent encore, bien sûr, dans ce domaine, tant les implications de l'adoption d'une monnaie unique sont nombreuses et complexes, mais ces mesures allaient dans le bon sens. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance est donc un texte important, qui enrichit le cadre de nos règles budgétaires. Né d'une crise grave, celle de la dette grecque, il place logiquement la discipline en vertu cardinale. Je ne dis pas que cet accord est parfait.

mettre en avant quelques idées simples. Avec l'euro, nous disposons de l'arme de souveraineté monétaire indispensable pour peser par rapport aux empires continents que j'ai cités tout à l'heure, à savoir les États-Unis, la Chine, et peut-être d'autres demain. Avec l'euro, et grâce à la politique de la BCE, nous permettons aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et à l'État français d'emprunter à des taux d'intérêt très peu élevés, il faut le dire.

laisser penser que, sans ce pacte de stabilité, nous pourrions dépenser sans compter, faire tourner la planche à billets, comme on disait autrefois, sans conséquence sur l'inflation, sans conséquence économique et sans conséquence sociale, c'est une blague

par le haut, bien sûr, et non pas par le bas. Mes chers collègues, dans mon bureau, il y a un seul portrait d'homme politique : celui de Robert Schuman, l'homme de la déclaration du 9 mai 1950. Aussi, je trouve heureux que, ici, au Sénat,

Le TSCG est un traité intergouvernemental, conclu en 2012 afin de renforcer les règles du pacte de stabilité et de croissance de 2001. Ce pacte stipule que le budget des États de la zone euro ne doit pas présenter un déficit supérieur à 3 % du PIB. De même, la dette publique ne doit pas être supérieure à 60 % du PIB de l'État. Ce pacte a été plusieurs fois complété, et c'est l'objet du TSCG. Ce dernier contient des règles budgétaires, dont celle de la limitation du déficit structurel des États parties au traité à 0,5 % de leur PIB. Le déficit structurel ne tient pas compte des effets conjoncturels de tel ou tel accident. Des aléas peuvent en effet toujours influer ponctuellement et temporairement sur les finances d'un État. C'est un progrès majeur. Mes chers collègues, rappelons-nous que le TSCG est un traité intergouvernemental. En clair, les vingt-cinq États qui en sont parties ont librement et contractuellement consenti aux obligations qu'il contient. Le TSCG n'a pas été imposé par Bruxelles Le débat d'aujourd'hui se fonde sur l'idée que le TSCG est caduc, puisqu'il n'a pas été transcrit dans le droit de l'Union dans le délai fixé à son article 16. l'obligation de transposition du TSCG dans le droit de l'Union n'était pas formulée à peine de nullité. Il se trouve, de source européenne, qu'une telle transposition est suspendue, mais pas annulée, par la commission du Parlement européen qui en a la charge. Au-delà de ces considérations, le groupe Les Indépendants considère que cette supposée caducité ne change pas grand-chose, et cela pour deux raisons. d'abord, les parties à ce traité ont volontairement souhaité son application. Ensuite, les dispositions du TSCG ont été inscrites dans les droits nationaux. La France a d'ailleurs procédé à cette inscription par le vote de la loi organique du 17 décembre 2012. Nous pensons cependant qu'il est possible et souhaitable de faire encore mieux. Le TSCG permet un déficit, si mineur soit-il. Nous souhaitons pour notre part qu'un budget ne puisse être voté qu'à condition qu'il soit excédentaire ou équilibré. Le véritable enjeu de ce débat sur la caducité du TSCG semble être ailleurs. Certains ont exprimé le sentiment que les États parties au TSCG, dont la France, ont été privés de leur autonomie budgétaire. Si l'on suit leur logique, retrouver cette autonomie ne signifierait rien d'autre que de pouvoir faire ce que nous nous sommes interdit : un déficit incontrôlé, voire incontrôlable. Les chantres du « dépenser plus en gagnant moins » rêvent peut-être, pour la France, de ce qui a conduit la Grèce et l'Europe au bord du gouffre

mais il s'agit d'une utopie dangereuse, qui enverrait le pays par le fond, comme elle l'a déjà fait pour un certain nombre d'autres États. Nous ne souhaitons pas une politique de dépense publique effrénée, parce qu'une telle politique mettrait en danger l'économie du pays et les avoirs des Français. Au contraire, nous sommes convaincus qu'il faut persister dans le choix de finances assainies, afin de fortifier notre économie et d'assurer l'indépendance de la Nation. De quelle autonomie budgétaire pourrait-il d'ailleurs être question, alors que la dette de la France atteint 98 % de son PIB ? Les Français dénonçaient déjà les excès de « Mme Déficit » voilà quelque deux Ils ont réaffirmé dernièrement qu'ils en avaient assez de l'irresponsabilité budgétaire. Nos concitoyens aspirent à ce que leur revenu et leur patrimoine ne soient pas dévalorisés par une gestion délirante du budget de l'État. Si, par extraordinaire, les obligations du TSCG venaient à tomber, au niveau tant national qu'international, le pacte de stabilité de 2001 continuerait à s'appliquer. Or lui aussi contient des mécanismes de sanction. Quand bien même nous serions entièrement autonomes sur la question budgétaire, faudrait-il que nous fassions n'importe quoi ? L'autonomie n'est pas la gabegie Les sanctions prévues par le TSCG visent à prévenir un danger bien plus redoutable : la sanction de l'Histoire. Tous ne le savent peut-être pas, mais, lorsque le chat n'est pas là, les souris ne sont pas obligées de danser. Elles peuvent choisir de travailler à préparer leur avenir ; elles peuvent choisir d'être responsables. Si nous respectons une saine gestion de nos finances publiques, ce n'est pas par peur des sanctions. C'est simplement le mieux que nous pouvons faire pour nos concitoyens et pour les générations à venir. Notre liberté, c'est aussi celle de nous engager. Or nous avons fait le choix de nous engager à assainir nos finances, et c'est tout à notre honneur. Contre le dangereux miroir aux alouettes d'une politique fondée sur le déficit, le groupe Les Indépendants continuera de promouvoir l'équilibre budgétaire. Il y va du sort de la France et de l'Europe. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, avant toute chose, je remercie le groupe CRCE de m'avoir fait rajeunir de quinze ans. En effet, j'ai eu l'impression, en préparant cette intervention, de me retrouver face à un sujet d'oral de concours. collègues, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas compris le sujet de la même manière que les orateurs précédents. Comme dans tout oral, je répondrai à cette question en trois parties, après m'être attardée quelques instants sur l'essence même du débat, à savoir la notion de caducité. En droit, un acte En droit, un acte juridique, régulier et valable lors de son édiction ou de sa création devient caduc dès lors que la survenance de certaines circonstances ou de certains faits l'empêche d'être exécuté. Il perd ainsi ses effets juridiques. L'anéantissement s'opère de plein droit du seul fait de la défaillance de la condition à laquelle il était soumis. La caducité résulte donc soit d'une condition qui était présente à l'origine, mais qui vient à disparaître ultérieurement, soit de la sanction d'une négligence, lorsqu'il incombait à une personne de réaliser une condition. La caducité est un acte extérieur à la volonté du législateur, qui s'impose à lui. Elle ne remet pas en cause la validité juridique du texte à l'origine, mais l'empêche de poursuivre ses effets. Avant de réfléchir sur les liens de cause à conséquence entre le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne, que vous me permettrez de désigner par l'abréviation TSCG, et l'autonomie budgétaire des États, il s'agit de vérifier que le postulat du groupe CRCE, à savoir la caducité dudit traité, est vérifié. Si tel est le cas, c'est que nous aurons répondu par l'affirmative à l'une de ces deux questions : une condition à l'origine du traité a-t-elle disparu ? ? Une négligence a-t-elle entraîné la non-réalisation de l'une des conditions ? Selon le premier paragraphe de l'article 1, le TSCG tend à « renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale ». De manière évidente, aucune condition à l'origine du traité n'a disparu, l'Union européenne n'a pas disparu et nous utilisons toujours des euros. Se trompant sur le sens juridique de la caducité, certains ont affirmé un peu vite la fin du TSCG devant l'incapacité de certains États signataires à respecter les règles fixées à l'article 3- un déficit structurel autorisé de 0,5 % pour l'objectif de moyen terme qu'à l'article 4 - une réduction d'un vingtième par an de l'écart entre la dette observée et la référence de 60 % du PIB. Moins de deux ans après son entrée en vigueur, force était de constater que l'Italie, le Portugal ou la Grèce avaient abandonné le chemin imposé de la réduction de leur dette. En France, le PLF pour 2015 reposait sur un déficit structurel de 2,2 %, soit le double du niveau fixé dans la loi de programmation budgétaire, loi d'application du traité. À l'époque, on n'envisageait pas un retour de la France dans le droit chemin avant 2019. Tel n'est malheureusement pas le cas. En effet, avant même les annonces du 10 décembre 2018 et celles du 25 avril 2019, le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis rendu sur le projet de budget pour 2019, soulignait que « les ajustements structurels prévus pour 2018- 0,1 point -et 2019- 0,3 point -, qui seront soumis à l'appréciation de la Commission, ne sont pas conformes aux règles du " bras préventif " du Pacte de stabilité Ce n'est pas parce que la France, sous François Hollande, comme sous Emmanuel Macron, ne réussit pas à s'astreindre à la rigueur budgétaire attendue que le TSCG devient inopérant pour autant. On peut simplement et malheureusement faire le constat de son inefficacité. C'est dans le titre VI, « Dispositions générales et finales », que nous pourrions trouver une négligence ayant entraîné la non-réalisation d'une des conditions. Comme l'a rappelé M. Laurent, l'article 16 précise que, dans un délai de cinq ans maximum à compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent traité doit être intégré dans le cadre juridique de l'Union européenne. La date butoir se trouvait donc fixée au 1 janvier 2018. À plusieurs reprises, les différentes instances européennes ont rappelé cet impératif : résolutions du Parlement européen des 12 décembre 2013 et 24 juin 2015 ; document de réflexion sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire présenté par la Commission en mai 2017 ; discours sur l'état de l'Union de 2017 proposition de directive du Conseil du 6 décembre 2017 établissant des dispositions en vue du renforcement de la responsabilité budgétaire et de l'orientation budgétaire à moyen terme dans les États membres. la résolution adoptée le 23 juin dernier par l'Assemblée nationale révèle que l'inscription du TSCG dans le droit de l'Union est loin d'être simple. On y lit notamment, au point 15 La proposition de la Commission européenne n'est pas consensuelle et son adoption est, aux yeux de certains États membres, compromise par d'importants obstacles juridiques ; [l'Assemblée nationale] invite, par conséquent, la Commission européenne à envisager des options alternatives pour renforcer le Mécanisme européen de stabilité dans l'hypothèse, fort probable, où l'unanimité exigée ne serait pas atteinte. » Ensuite, au point 16, l'Assemblée nationale « considère, dans cette perspective, que le renforcement du Mécanisme européen de stabilité pourrait se faire une révision du traité intergouvernemental qui l'instaure et souhaite qu'une réflexion soit engagée pour doter ce mécanisme d'instruments et de pouvoirs préventifs de gestion des crises ». La non-réalisation de son article 16 fait-elle tomber le TSCG ? C'est la lecture faite par M. Mélenchon, et que partage M. Laurent. Ce n'est pas la mienne. Il me semble que la non-réalisation de l'article 16 est surtout révélatrice des difficultés de la construction européenne, notamment sur le plan économique, dans un contexte de croissance économique

et si chaque pays de l'Union avait des politiques budgétaires irresponsables, nous serions bien vite rattrapés par un principe de réalité : la réalité des marchés. C'est déjà le cas ! Les règles du TSCG sont là pour protéger la zone euro et non pas pour la livrer aux marchés, voire au FMI.

quelle serait la liberté d'un pays asphyxié par la dette ou soumis à l'hyperinflation ? Les exemples contemporains nous montrent qu'un mauvais TSCG vaut mieux qu'un défaut de paiement sur la dette. Il faut conclure, ma chère collègue. La Grèce n'a pas sombré ; le Venezuela ne peut pas en dire autant

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je rends hommage à la leçon de droit

? Je ne le pense pas non plus. Selon moi, nos dépenses publiques, dont la maîtrise passe non par des coupes brutales, mais par le ralentissement de leur croissance en volume, évoluent conformément aux engagements que nous avions pris. On voit d'ailleurs que nous ne sommes pas dans une période d'austérité budgétaire. Les résultats sont, en revanche, plutôt positifs. En effet, nous avons créé 600 000 emplois en deux ans, et les investissements productifs

L'économiste Jean Pisani-Ferry déplore que l'objectif d'un déficit structurel à zéro empêche les gouvernements de profiter des taux d'intérêt durablement bas, qui sont ceux d'aujourd'hui,

Un certain nombre d'économistes allemands et français ont proposé de substituer aux règles actuelles une règle unique fondée sur le taux de croissance des dépenses publiques.

émettent, dans un certain nombre de cas, ce qu'on appelle des « obligations juniors », c'est-à-dire dont le degré d'appel est moins important que les autres éléments de l'actif. Enfin, le vrai débat porte sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Nous avons proposé la mise en place d'une union budgétaire reposant non seulement sur la surveillance des politiques budgétaires nationales, mais aussi sur la solidarité. Le ministre passe Le ministre passe beaucoup de temps à essayer de convaincre ses partenaires. L'Allemagne semble avoir évolué de façon positive, acceptant le principe de la création d'un budget pour la zone euro, qui permettrait aux États membres de financer les investissements d'avenir et de mieux résister aux chocs macroéconomiques.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a maintenant plus de sept ans, le 2 mars 2012, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union européenne a été signé. Par ce traité, vingt-cinq des vingt-huit États membres de l'Union européenne se sont engagés, et engagés librement, de manière souveraine, à respecter des règles de discipline budgétaire.

Je reviendrai sur ces deux concepts un peu plus tard, car il convient, avant tout, de rappeler quels ont été les germes de ce traité et quelles en sont les ambitions. Le TSCG entend astreindre les États de la zone euro qui en sont signataires à financer leurs dépenses par leurs recettes, afin de limiter le recours à l'emprunt.

et que nous connaissons, les États membres ne sont pas parvenus à respecter les règles strictes prévues par le pacte de stabilité et de croissance adopté en 1997 en vue de la création de l'euro, le 1 janvier 1999. Ils se sont livrés à des excès d'endettement et de déficits préjudiciables à l'ensemble de la zone euro, outrepassant, somme toute, la limite des 3 % de déficit autorisé et ce, plusieurs années durant. Aussi, en 2011, ce nouveau traité est venu proposer des règles communes de gouvernance économique et budgétaire, afin de veiller à ce que les pays soient contraints de s'astreindre à une certaine discipline budgétaire. Le TSCG prévoit également une coordination et une convergence des politiques économiques. Les États concernés sont tenus de communiquer leurs plans nationaux d'émissions de dette publique et de s'assurer que les grandes réformes économiques qu'ils entendent réaliser sont débattues au préalable et, au besoin, coordonnées. Par conséquent, en son article 1, le TSCG prévoit logiquement que les parties contractantes « conviennent, en tant qu'États membres de l'Union européenne, de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d'un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière de croissance durable, d'emploi, de compétitivité et de cohésion sociale En contrepartie d'une solidarité financière, le pacte budgétaire européen introduit une règle d'or, qui engage les États signataires à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit « en équilibre ou en excédent

Cette responsabilité est indispensable, car chacun sait que l'un des risques majeurs de la zone euro est de voir poindre des politiques budgétaires tout à fait insoutenables. La discipline est indispensable au fonctionnement de l'Union européenne., vouloir s'extraire du TSCG, c'est avant tout prendre le risque d'ouvrir la porte à des politiques budgétaires insoutenables et, à terme, à l'implosion des banques, à une nouvelle crise économique et à l'explosion de la zone euro. Voilà le véritable risque et l'enjeu qui nous occupe ! En outre, ces règles économiques ne tombent pas du ciel. Il ne s'agit pas d'un artefact créé de toutes pièces. Au-delà des notions de discipline et de sérieux économique, indépendamment du contexte dans lequel elles sont apparues, ces règles ont une raison d'être en elles-mêmes, à savoir l'interdépendance entre les États membres. Nous sommes liés les uns aux autres, que nous le voulions ou non ; et, en l'espèce, nous le voulons. En effet, quand bien même les règles du TSCG seraient caduques, les marchés financiers viendraient nous rappeler, sans doute douloureusement, à cette réalité de l'interdépendance entre les États. Enfin, présenter le TSCG comme un carcan ou un instrument de servitude obligeant les États à s'appliquer une austérité permanente et généralisée n'est pas conforme à la réalité de ce traité.

Permettez-moi, à ce titre, de souligner que les notions de TSCG et de politique budgétaire expansionniste ne sont pas incompatibles. Le TSCG oblige à l'équilibre ; il ne condamne pas à l'austérité.

ce qu'ils considèrent comme le dogme de l'austérité, je rappelle que les dérives budgétaires nationales créent des crises, et qu'il nous incombe à tous de faire preuve d'intelligence budgétaire et de responsabilité. C'est à cette responsabilité que nous rappelle le TSCG. La parole

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord remercier tous les orateurs qui sont intervenus dans ce débat de la qualité de leurs interventions : M. Leconte, du rappel historique des différents engagements pris par la France sur la scène européenne avec ses partenaires

Nous estimons que les États parties au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance ont choisi, en mars 2012, et en pleine indépendance, au-delà des avis exprimés alors par telle ou telle force politique de leurs pays respectifs, de signer ce traité, car il leur a semblé que cela répondait à leurs intérêts. Il ne s'agissait en aucun cas de renoncer à notre souveraineté budgétaire- laquelle est pleinement exercée par le Parlement -, mais bien de coordonner nos décisions au sein de la zone euro. Au sein de celle-ci, la coordination des politiques budgétaires nous paraît essentielle. La politique budgétaire d'un pays a des conséquences sur tous les autres membres de l'union monétaire. Un pays qui a sa propre monnaie ne peut pas faire ce qu'il veut sur le plan budgétaire, car il est très vite rattrapé par l'évolution de sa monnaie, laquelle agit comme une corde de rappel très forte. Nous avons connu cela à de nombreux moments, avec le franc au début des années 1980 et encore en 1992 et 1993. Désormais, l'union monétaire nous en protège, avec avec comme contrepartie la nécessité d'éviter des comportements désordonnés ou non coopératifs. La convergence des taux d'intérêt au sein de la zone euro nous permet de nous endetter à bas coût. C'est évidemment un autre avantage souligné par beaucoup d'entre vous. savons, c'est-à-dire que si un pays abuse de cette possibilité, il peut provoquer une crise globale de la zone euro, laquelle peut se déclencher brutalement, en suscitant une instabilité financière dans toute la zone monétaire, comme ce fut le cas lors de la crise grecque. Les règles budgétaires communes représentent, de ce point de vue et selon nous, une protection pour tous les États. Ce cadre commun dont nous nous sommes dotés est aussi utile sur le plan strictement national. En effet, peut-être l'aurions-nous fait indépendamment de notre engagement, mais force est de constater que ce traité nous a conduits à renforcer notre Haut Conseil des finances publiques, le HCFP, et notre programmation pluriannuelle des finances publiques. Cela donne ainsi plus de crédibilité et de vision à moyen terme sur nos comptes publics. Cela participe pleinement du bon fonctionnement de notre démocratie, car le Parlement peut se prononcer en connaissance de cause sur la base d'informations solides et transparentes. De plus, la logique du traité, qui consiste à maîtriser la dette publique, mais en tenant compte de la situation économique, est efficace. Nous devons faire plus d'efforts quand la croissance est bonne, mais aussi pouvoir relâcher la contrainte en cas de ralentissement marqué de la conjoncture économique. C'est précisément ce que vise le TSCG, qui repose sur des objectifs calculés en « structurel La question qui se pose à travers votre débat demandé par le groupe CRCE, et que j'ai entendue dans certaines de vos interventions, est la suivante : quelle politique budgétaire devrait être

Les mesures que le Gouvernement a prises récemment en sont l'exemple ou la démonstration. Nous conservons une large capacité d'action au niveau national pour tenir compte des circonstances propres à notre situation. Ainsi, la politique que nous conduisons montre que nous pouvons nous adapter, tout en visant notre objectif de réduction de la dette. Notre stratégie budgétaire de tenue des comptes publics et de baisse de la dette a été définie d'abord parce qu'elle est, à nos yeux, bonne pour notre pays, et non pas eu égard au traité qui nous engage. Nous considérons- je sais que beaucoup ici partagent cette idée -qu'une dette trop élevée est néfaste pour nos concitoyens, et cela pour au moins trois raisons. Tout d'abord, les dépenses afférant au service de la dette sont autant d'argent public qui pourrait servir au financement des services publics ou à des investissements favorables à la croissance de long terme. Ensuite, une dette trop élevée peut conduire à une perte de souveraineté si la confiance des marchés n'est plus là.

Nous serions dans la main des investisseurs, ce que nous ne souhaitons pas. Enfin, au risque d'énoncer une évidence, une dette trop élevée est un fardeau pour les générations futures. Nous ne voulons pas laisser à nos enfants la charge des dépenses que nous faisons aujourd'hui. Mesdames, messieurs les sénateurs, je suis, comme nombre d'entre vous, un élu local. J'ai été maire de ma commune pendant près de dix ans et, comme tous les élus locaux, je sais- et nous savons tous -que si nous ne maîtrisons pas nos comptes publics, nous nous privons de toute marge de manoeuvre en cas de crise ou tout simplement en cas de besoin. Je l'ai fait dans ma propre commune, en réduisant les dépenses de fonctionnement sans remettre en cause la qualité des services rendus- ceux-ci ont même été renforcés. Je l'ai fait aussi en réduisant de moitié la dette, tout en augmentant très fortement les investissements. Cette expérience n'est pas isolée, je le sais, et je crois que, traité ou non, nous sommes nombreux à former le voeu d'une situation identique pour les comptes nationaux. En conclusion, pour revenir à notre débat national et européen d'aujourd'hui, le Gouvernement que je représente devant vous porte la conviction qu'une stratégie de réduction de l'endettement public est une stratégie de protection de l'autonomie budgétaire du pays. J'ai en tête des exemples récents, tel celui de l'Italie, dont la charge d'intérêt est si élevée que le poids de sa dette croît mécaniquement, en dépit d'excédents budgétaires primaires hors charge d'intérêt, et qui, sous la pression d'une montée des taux d'intérêt, a dû amender substantiellement sa stratégie budgétaire. Par ailleurs, nous considérons que la stratégie de réduction du déficit et de la dette choisie par le Gouvernement nous permet d'endiguer la hausse constante de la dette grâce aux efforts budgétaires que nous déployons quotidiennement. Notre cap reste celui d'une réduction de l'endettement et du déficit d'ici à la fin du quinquennat.

Cette réduction de la dette et du déficit passe par un effort sur la dépense publique en ciblant les endroits où des économies sont possibles, notamment grâce aux nouveaux outils digitaux, mais pas seulement. Ces efforts ne doivent pas se faire au détriment des investissements publics qui sont essentiels à la croissance de long terme et donc à la soutenabilité des finances publiques- c'est là le rôle du grand plan d'investissement.

Il nous faut appliquer un nouveau modèle budgétaire : moins de dépenses publiques et de dette, moins de prélèvements obligatoires, mais plus de soutien à l'investissement et à l'innovation. Notre objectif reste de réduire le poids des dépenses publiques de près de 3 points en équivalent PIB sur le quinquennat et de réduire de plus de 1 point Au-delà des efforts de consolidation budgétaire, une stratégie de renforcement des finances publiques doit aussi s'appuyer sur des leviers de renforcement de la croissance et de l'efficacité de l'action publique. La baisse des dépenses publiques doit donc aller de pair avec des réformes structurelles. Il faut attaquer les problèmes sociaux à la racine, plutôt que de traiter systématiquement leurs symptômes.

De ce point de vue, je le répète, le traité de 2012 ne nous empêche nullement de conduire la politique budgétaire qui nous semble la plus adaptée pour la France. Au contraire, il nous a permis de renforcer notre cadre budgétaire pour plus de transparence et, finalement, de donner plus de crédibilité à nos comptes publics. Il nous permet aussi, et peut-être surtout,